Vous le savez, depuis sa mise en oeuvre, nous n'avons cessé de dénoncer une mesure inefficace. Force est de constater que nous avions raison : la n'a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française. J'en veux pour preuve un rapport récent de France Stratégie indiquant que les gains fiscaux issus de la création de la en 2018 se sont concentrés sur les ménages les plus aisés. Les dividendes perçus ont ainsi crû de 62 %, soit 9 milliards d'euros, sachant que

est une fantaisie ; deuxièmement, la seule mesure ayant permis de faire progresser le pouvoir d'achat des Français a vu son coût acquitté par ces mêmes Français : ceux qui ne paient plus la taxe d'habitation paient quand même, la réduction forcée de la voilure d'action des collectivités territoriales, en difficulté financière. Si l'on prend en compte l'ensemble de la politique fiscale du Gouvernement, les 10 % de ménages les plus aisés ont profité de 79 % du gain total de niveau de vie.

». Toutefois, la situation est loin d'être aussi idyllique. En effet, cette hausse des dividendes s'est faite au détriment des autres usages des profits, à savoir l'investissement et la rémunération des salariés. Le taux d'augmentation de l'investissement des sociétés non financières est passé de 5 à 3,9 %.

Je note en outre que le PFU a permis de rapprocher le régime fiscal français de celui d'un grand nombre de nos partenaires européens.

clairement établi que la « barémisation » des revenus du capital, en 2013, s'était en réalité traduite par une contraction de la base fiscale, et avait d'ailleurs

qui permet de se faire payer en dividendes et non pas en salaires. Dans certaines tranches de revenus, vous avez objectivement intérêt à vous faire verser des dividendes et pas des salaires. salaires. On sait depuis de très longues années que le capital est moins imposé que les salaires, que le partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les revenus du capital est défavorable au monde salarié.

cette question du financement de la dette publique allait se poser. Il faut donc peut-être d'ores et déjà commencer à faire en sorte que ceux qui ont la capacité de contribuer un peu plus contribuent un peu plus. D'où l'idée de supprimer l'abattement de 40 % qui s'applique aux dividendes pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La

pour l'imposition des dividendes que lorsque s'applique le barème de l'impôt sur le revenu. Depuis 2018, lorsque le contribuable n'opte pas pour l'imposition au barème, les dividendes sont imposés au PFU et l'abattement de 40 % n'est plus appliqué. Par conséquent, la suppression de l'abattement pénaliserait avant tout les contribuables qui optent pour l'imposition au barème, donc,, les moins aisés.

Cette proposition avait d'abord été formulée par les membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat, avant d'être écartée au titre des fameux « jokers » du Président de la République. Elle vise à instaurer une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes. Outre les ressources supplémentaires qu'elle permettrait de dégager afin d'amoindrir les effets économiques de la crise sanitaire, une telle taxe permettrait d'encourager le déploiement des bénéfices des entreprises en direction des investissements d'avenir et des emplois. Quel est l'avis de la commission Je vais proposer que les élus de notre assemblée, élus au suffrage indirect de second degré, répondent à une proposition des membres tirés au sort

par les entreprises, je ne souscris pas à cette proposition. J'émets donc un avis défavorable

sont malins la plupart des patrons de ces très grands groupes qui versent des dividendes ? Ils se paient sous forme d'actions, et ils mènent une politique d'entreprise favorable aux actionnaires en se versant de plus en plus de dividendes

Je veux dire à mes collègues que j'ai beaucoup de respect pour les femmes et les hommes qui sont engagés dans des démarches participatives. Ne déformez pas mes propos ! J'ai simplement dit qu'une assemblée parlementaire répondait

amendement vise à rétablir le système d'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. Ce régime a été réformé, et on a supprimé le dispositif anti-abus en réduisant le délai de détention des plus-values

vise à renforcer la contribution des ménages les plus aisés à la solidarité nationale en rehaussant le taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. À la différence de l'amendement précédent, les deux taux considérés

Le produit de ce surcroît pourrait atteindre 2 milliards d'euros, qui seraient les bienvenus en cette période d'écroulement des recettes de l'État. Un tel dispositif réintroduirait de la justice fiscale et sociale.

2020, une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises, dont nous avons beaucoup parlé, et surtout des ménages en difficulté. Le présent amendement vise à mettre en place un prélèvement exceptionnel et unique de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale. nationale. Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d'assurance vie supérieurs ou égaux à 150 000 euros, par référence aux dispositions déjà existantes en matière d'assurance vie.

s'est révélée n'être qu'une quasi-privatisation de l'épargne populaire. Douze ans après la mise en oeuvre de cette réforme, il apparaît que la fin du monopole de distribution du livret A par les caisses d'épargne et La Poste s'est en réalité muée en privatisation de l'épargne

appuyer l'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, la transition agroécologique ou encore le déploiement d'une politique préventive de santé publique centrée sur l'alimentation.

? Ces amendements visent à prévoir, dans les mêmes zones que le « Denormandie ancien » et selon des modalités différentes, une réduction d'impôt pour l'acquisition d'un local commercial neuf ou faisant l'objet de travaux.

arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il semble que le Gouvernement n'ait pas l'intention de le proroger. Or ce crédit d'impôt accompagne les personnes qui financent l'installation d'équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d'améliorer l'adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes. Le Président de la République n'avait-il pas pris l'engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ? Le Gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte d'effectuer les travaux d'adaptabilité ; rien n'est fait pour les accompagner et leur simplifier l'accès au logement. Par ailleurs, compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population et de l'objectif de donner à chacun la possibilité de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile, il est proposé de proroger la période d'application de ce crédit d'impôt sur le revenu pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Il est également proposé d'actualiser les plafonds de travaux qui peuvent donner lieu à crédits d'impôt, ces plafonds n'ayant jamais été actualisés depuis 2005.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que plus de 7 millions de Français éprouvent des difficultés à assumer le premier poste de dépenses des ménages, le logement. Certains bailleurs sociaux parlent déjà de 10 % de loyers impayés depuis le début du confinement, mais le risque majeur de défaut de paiement de loyer et de charges est encore devant nous, avec, à terme, la menace d'expulsions. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la structure du logement en France. Le Centre de recherche

dans la petite couronne, vous constaterez que le taux de vacance des bureaux commence à être significatif, notamment à La Défense.

ne me semble pas approprié de priver ce réseau de ces financements, alors même que les transports en commun souffrent d'importantes pertes de revenus, à Paris comme ailleurs.

En outre, l'investissement dans un fonds de logement n'est pas aussi risqué que l'investissement dans un fonds commun de placement à risque (FCPR), dont vous souhaitez emprunter le régime fiscal en exonérant les plus-values des cessions de parts après cinq ans de détention.

Dans mon département des Hauts-de-Seine, confronté à une demande criante, récurrente, énorme de logements, il serait inconcevable de laisser des tours à moitié

drastiques de confinement mises en place et de l'interruption des flux touristiques. Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d'emplois à la clé. Les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les prêts garantis par l'État souscrits par les professionnels vont devoir commencer à être remboursés, alors même que la situation économique des entreprises est encore plus fragile, après des mois de graves difficultés et aucune perspective de reprise dans les mois à venir. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie prévoit que le retour à une activité normale prendra plusieurs années. Face à cette situation, les hôteliers font preuve d'initiative et se réinventent pour ne pas sombrer, en proposant de nouvelles activités, notamment la transformation de chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs. Afin de soutenir cette filière qui se bat pour survivre, cet amendement tend à prévoir que les entreprises du secteur de l'hôtellerie particulièrement touchées par la crise pourront bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France. Tel est l'objet du présent amendement.

tend à exclure des surfaces taxables pour le calcul de la taxe à usage de bureaux les seuls emplacements équipés d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Une mesure incitative de cette nature est nécessaire, compte tenu des coûts d'installation et de fonctionnement des bornes dans ces ouvrages. Celles-ci engendrent des frais élevés de raccordement et de mise aux normes de sécurité incendie, ainsi que des frais de maintenance et d'entretien. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

et, pour tout vous dire, je ne vois pas de raison décisive d'accepter cette exonération au regard de l'objectif de la taxe, qui est de financer certains organismes, et non

Le fait de rendre déductibles ces agrandissements inciterait davantage les bailleurs privés à engager des rénovations dans leurs propriétés, ce qui permettrait de lutter contre les logements vacants. Quel Pour éviter tout quiproquo, je veux rappeler le droit existant. L'article 31 du code général des impôts prévoit que les dépenses d'amélioration des logements sont déductibles des revenus fonciers, sauf lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. L'amendement tend à inclure les travaux d'agrandissement parmi les dépenses d'amélioration déductibles du revenu net.

Ce déficit peut être imputé sur le revenu global du contribuable et réduire ainsi son imposition, dans la limite d'un plafond fixé à 10 700 euros. C'est un outil apprécié des bailleurs et un mécanisme vertueux. Il favorise la mise en location sur longue durée de biens immobiliers entretenus, puisque seules sont éligibles les dépenses liées à des travaux de réparation et d'entretien, c'est-à-dire des travaux au service immédiat des locataires. Le plafond du déficit foncier n'a pas été révisé depuis la loi de finances pour 1995. Or engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût bien supérieur aux dépenses d'entretien usuelles. Il serait donc souhaitable d'utiliser ce dispositif pour encourager les propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux, en cohérence avec le plan de relance et l'urgence écologique. Depuis six ans, malgré l'enjeu environnemental de la rénovation énergétique des bâtiments, les bailleurs n'ont pas bénéficié des dispositifs d'accompagnement de la rénovation énergétique et ont donc délaissé ces travaux trop coûteux. coûteux. Le fait de ne pas avoir engagé ces travaux de rénovation s'exerce partout au détriment des locataires, mais, en copropriété, cette situation est doublement pénalisante, à la fois pour le locataire et pour l'ensemble de l'immeuble. Faute de moyens ou d'accompagnement, les copropriétaires-bailleurs n'ont en effet pas été enclins à voter les travaux nécessaires pour toute la copropriété. Cet amendement vise donc à doubler le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu'une part significative- 40 % -du montant des travaux est composée de travaux d'économie d'énergie, d'énergie, collectifs ou individuels. Il s'agit de mettre en cohérence ce dispositif vertueux avec la réalité du coût des travaux de rénovation énergétique. Pour éviter tout effet d'aubaine, les propriétaires bailleurs ayant recours à ce doublement du plafond du déficit foncier perdraient le bénéfice de MaPrimeRénov'pour

Elle contribue à un partage plus équitable des richesses, en rapprochant les intérêts des employés de ceux des employeurs. Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l'avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C'est pourquoi il convient d'en renforcer l'attractivité, notamment auprès des entreprises. Jusqu'en 2012, l'un des intérêts de la participation, pour les entreprises, résidait dans la constitution d'une provision pour investissement qui ouvrait droit à un avantage fiscal important. Ce mécanisme a été supprimé en 2012. Le présent amendement vise à le rétablir, afin de renforcer l'attractivité de la participation pour les entreprises. Quel est l'avis de la commission ? J'émets un avis

quand cette provision était encore déductible de l'impôt sur les sociétés, montrent que cette dépense fiscale est en fait assez peu efficace.

Le code de commerce prévoit une neutralité des opérations d'apport d'actions gratuites par les salariés à une société ou en cas d'opération de restructuration. Dans ce cas, l'opération est sans incidence sur le régime des actions gratuites accordées aux salariés. Le second alinéa du III de l'article 80 du code général des impôts reconnaît la même neutralité de ces opérations, mais ajoute trois conditions, dont celle, visée par cet amendement, de l'ouverture à l'ensemble des salariés, qui s'est avérée bloquante pour la diffusion du mécanisme d'actions gratuites à un grand nombre de salariés. Or la perspective de ne pouvoir rassembler les actions dans une holding commune est dissuasive, notamment pour les sociétés non cotées. Afin de s'assurer du développement des opérations d'actionnariat salarié dans le plus grand nombre d'entreprises, notamment dans des entreprises de petite taille, cet amendement vise à supprimer cette condition.

dans des conditions précises qui garantissent que l'opération contribue bien à l'objectif visé, notamment l'obligation d'attribuer des actions gratuites à l'ensemble des salariés. À l'inverse, la disposition que vous proposez, en supprimant cette condition, pourrait accorder un avantage sans justification à des dirigeants qui souhaiteraient reprendre la société émettrice au moyen d'une holding dédiée. Cette disposition serait donc en contradiction avec l'objectif affiché de développement des opérations d'actionnariat salarié pour le plus grand nombre. Madame Vermeillet, l'amendement

quel que soit leur nombre, dès lors que la société de gestion est bien entendu en mesure de retracer le respect du quota fiscal. De plus, ce dispositif permet d'harmoniser les règles françaises avec celles en vigueur pour la concurrence étrangère

En cas de multiplication des niveaux d'interposition entre les porteurs de parts et les sociétés bénéficiaires, le risque est dilué et l'avantage perd sa justification. L'absence de limitation de niveau d'interposition pour le calcul du quota fiscal rend difficile en pratique le contrôle de ce quota- voilà une première raison qui explique notre opposition à la disposition que vous proposez. Par ailleurs, cette absence de limite pourrait aboutir à une situation paradoxale, où le quota fiscal du code général des impôts serait plus favorable que le quota juridique du code monétaire et financier prévu pour les FCPR. Pour ces deux raisons,

prévu par l'article 117 du code général des impôts constitue un acompte d'impôt sur le revenu : il n'a pas vocation à être appliqué à des revenus exonérés d'impôt sur le revenu. Les dividendes perçus dans le cadre d'un plan d'épargne retraite (PER) sont exonérés d'impôt sur le revenu, comme l'ensemble des revenus détenus dans les plans d'épargne salariale et les plans d'épargne retraite visés à l'article 163 B du code général des impôts. Cet amendement vise à ne pas amputer les dividendes versés dans un PER du prélèvement du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être,, remboursé à l'épargnant, car ces dividendes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Faire peser sur l'épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable ne favorise pas le développement du PER compte-titres, qui a constitué une des principales innovations du nouveau PER. En effet, la perception en amont du prélèvement diminuera le rendement du PER compte-titres et son attrait par rapport au mais impliquera nécessairement une procédure de récupération selon des modalités qui ne sont pas connues, puisque l'impôt n'est pas dû. Il est, en outre, difficile d'expliquer les raisons d'une différence de traitement fiscal entre, d'une part, les intérêts issus d'un PER et les dividendes issus de titres détenus d'un PEA, qui sont dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire et, d'autre part, les dividendes issus d'un PER, alors que ces revenus sont tous exonérés d'impôt sur le revenu lors de l'imposition définitive. Quel

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement n'est pas opposé en soi à un lissage du traitement fiscal applicable aux produits d'épargne qui bénéficient de la même exonération d'impôt sur le revenu. La proposition présentée par Mme Vermeillet rappelle à juste titre que le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux dividendes versés dans un PER, dès lors que ces mêmes dividendes sont exonérés d'impôt sur le revenu, s'ils sont réemployés dans le plan et donc frappés d'indisponibilité. Cependant, votre proposition mérite d'être expertisée plus avant, pour s'assurer de sa portée et de son exhaustivité, en lien notamment avec les organismes gestionnaires des PER, qui sont chargés du recouvrement des prélèvements. Il serait fâcheux que, malgré la bonne intention que nous partageons, elle puisse engendrer des difficultés, par une interprétation, pour d'autres dispositifs proches du PER, qui ne seraient pas expressément cités dans le texte- je pense notamment au régime fiscal du plan d'épargne entreprise. Il est donc souhaitable de clarifier

La loi Pacte du 23 mai 2019 avait notamment pour ambition de rendre plus attractif le régime de l'épargne retraite. Les débuts du plan d'épargne retraite individuel semblent encourageants. Pour maintenir et conforter cette attractivité du plan d'épargne retraite, il semble aujourd'hui nécessaire de prévoir l'exonération des plus-values immobilières réalisées, à travers un PER compte-titres, sur les parts de sociétés Celles-ci peuvent être placées sur un PER individuel pouvant donner lieu à l'ouverture d'un compte-titres, disposition créée par la loi Pacte du 23 mai 2019. En outre, afin de préserver le rendement de l'épargne retraite placée sur le PER, il est souhaitable de prévoir une telle exonération, afin d'aligner le traitement fiscal des plus-values immobilières sur celui des plus-values mobilières et de ne pas créer de dichotomie de traitement fiscal entre ces deux types de plus-values. Dans le cas contraire, cela dissuaderait l'épargnant d'investir dans de telles parts. À cet effet, il convient de créer un article 150 UE du code général des impôts, objet du présent amendement. Quel est l'avis de la commission ? J'oppose un avis

L'article 163 du code général des impôts prévoit déjà que les revenus des titres détenus dans un PER sont exonérés, s'ils sont réemployés dans le plan, sans distinction selon la nature du titre.

d'une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 euros tous les quinze ans ; d'autre part, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. De nombreux facteurs justifient de fluidifier la circulation du capital par l'assouplissement des conditions pesant sur les donations. Je pense notamment à l'allongement de la vie, à la très forte concentration du capital dans les populations âgées et aux inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser. Je vous propose donc, d'une part, de porter la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d'autre part, de supprimer la condition d'âge maximale pour le donateur, fixée aujourd'hui à 80 ans.

Ce chiffrage donne une idée du coût de l'amendement, si nous réduisions de sept ans le délai de rappel fiscal pour l'ensemble des donations. Je rappelle également que l'exonération temporaire à hauteur de 100 000 euros, sous condition de réemploi, a déjà été introduite sur l'initiative du Sénat, dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative de cette année. Il faut raison garder sur ce dispositif, et privilégier des dispositifs qui seraient plus susceptibles de soutenir la reprise.

le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit, quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux. Il vise tout à la fois la simplification et l'équité, en instaurant un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.

La définition d'une progressivité plus linéaire, autour d'un montant pivot fixé à 350 000 euros, semble plus équilibrée. Il s'agit de l'application de la volonté de lissage et de hausse de la progressivité de la fiscalité de la transmission du patrimoine, qui demeure aujourd'hui particulièrement discriminante. Nous proposons de créer des seuils de 15 000, 30 000, 60 000, 180 000, 460 000 et 720 000 euros, afin de lisser la progressivité réelle de l'imposition. Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Nous estimons que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 euros seront globalement moins taxées, quand celles percevant quand celles percevant une succession supérieure à 350 000 euros le seront davantage, l'impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas. Ce seuil ne peut que sembler très raisonnable et ne pénalisera en aucun cas la classe moyenne ; il ne concernera que les successions les plus importantes. Il convient également d'ajouter

commission ? Je demande le retrait de l'amendement de M. Delahaye. Les transmissions en ligne indirecte représentent plus de la moitié des recettes des droits de mutation à titre gratuit, contre seulement 10 % des montants transmis. Il n'est donc pas illégitime de maintenir une imposition différenciée selon le lien de parenté, dès lors que cela encourage les transmissions familiales.

rapprocher les dates au cours desquelles des donations peuvent être faites, à tel point que vous proposiez de permettre la donation de 150 000 euros par enfant et par parent tous les dix ans, qui représente des montants sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. Entre octobre 2019, où vous souhaitiez alléger très fortement les droits de mutation sur les donations, et aujourd'hui, où vous nous proposez de les renforcer, j'ai du mal à m'expliquer ce revirement.

une disposition prise en 2012, puisque la majorité socialiste a augmenté les droits de donation et de succession pour les familles, en diminuant à 100 000 euros l'abattement pour les transmissions en ligne directe. Le présent amendement propose de revenir au, en ramenant cet abattement à 159 325 euros.

en effet nécessaire d'adapter les DMTG à l'allongement de l'espérance de vie et à l'évolution des relations familiales et sociales. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir,

à faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin. Quel Je demande le retrait de ces deux amendements, parce que, comme je viens de le dire, nous ne souhaitons pas modifier le dispositif que nous avons adopté ici lors de l'examen de la troisième loi de finances rectificative.

Il est ainsi proposé d'insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires-héritiers ayant revendiqué l'application d'un pacte d'engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel complémentaire de conservation des titres pour une durée de quatre ans débutant à l'issue de l'engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil. Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d'une exonération partielle de 90 %.

c'est le fameux pari des entreprises de long terme. Ce dispositif extrêmement puissant permet de s'assurer que les entreprises françaises demeurent dans le giron national. Je vous propose un

constitutionnel. En effet, un taux d'exonération de 90 % pourrait être jugé excessif, même si l'interdiction de cumuler cette exonération bonifiée avec la réduction d'impôt pour âge du donateur constitue en quelque sorte un gage de sécurité.

Afin de favoriser l'implication des salariés dans la vie des entreprises, notamment les plus petites, il est proposé d'étendre ce dispositif aux donations de parts sociales et de titres, sachant que ces donations sont limitées à 15 % du capital de l'entreprise et que les parts ou actions concernées doivent être détenues depuis deux ans. Ce dispositif va dans le sens du partage de la valeur des entreprises, tel que l'a voulu la loi Pacte, en développant l'actionnariat salarié. Il lève un frein, en élargissant le régime existant prévu à l'article 790 A du code général des impôts. Quel Je partage la volonté d'encourager les donations d'entreprises aux salariés, mais je veux soulever deux problèmes importants. contrairement aux dispositifs qui existent pour les fonds de commerce et les entreprises individuelles, l'exonération prévue dans cet amendement n'est pas plafonnée à 300 000 euros. part, cette exonération n'est subordonnée à aucune condition de poursuite de l'activité par les repreneurs, alors que, pour le dispositif applicable aux fonds de commerce, les donataires doivent rester à la tête de l'entreprise pendant au moins cinq ans.

de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces, lorsque ces sommes sont notamment affectées, dans les trois mois, à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne. Toutefois, en limitant le bénéfice du dispositif aux seules entreprises de moins de cinquante salariés, donc en excluant les PME, et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons éligibles, alors même que le montant moyen des prêts garantis par l'État s'élevait déjà à 135 000 euros

En effet, pour pouvoir entrer en vigueur immédiatement, le dispositif d'exonération temporaire qui a été introduit cet été sur l'initiative du Sénat a été placé sous un régime d'exemption réservé aux petites entreprises qui sont les plus concernées par les difficultés d'accès aux financements.

neveu ou nièce à défaut -, dans la limite de 100 000 euros et à la condition que la donation soit affectée à la construction de la résidence principale. Il existe cependant une ambiguïté : est-ce que l'acquisition d'un logement neuf en vente

à M. Guillaume Gontard. Le Gouvernement a introduit une exonération de dons pour les enfants et les petits-enfants, et ce jusqu'à 100 000 euros.

les 10 % des ménages les mieux dotés possèdent au minimum un patrimoine de 534 800 euros, alors que les 10 % les plus modestes détiennent au maximum un patrimoine de 3 000 euros, soit pratiquement deux cents fois moins.

le cadre de l'examen de la troisième loi de finances rectificative qui vise à encourager les Français à réinjecter leur épargne dans l'économie réelle.